Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a sollicité ce débat sur la situation des urgences durant l’été 2024 afin de prendre la mesure des difficultés structurelles qui affectent notre système de santé et de demander au Gouvernement comment il compte assurer une bonne prise en charge aux urgences pour tous et partout sur le territoire.

Il ne s’agit pas d’une question technique. Derrière chaque chiffre se trouve une réalité douloureuse : des patients laissés de longues heures sur des brancards ou dans des véhicules de secours, emmenés d’un hôpital à l’autre, des soignants épuisés ne pouvant pas prendre leurs congés, des services en tension permanente.

sur un brancard. C’est indigne de notre système de santé, de notre service public et de notre République ! L’arrêté du 2 juillet 2024 relatif à la régulation temporaire de l’accès aux urgences n’apporte qu’une solution transitoire et partielle.

La mission Braun avait pourtant esquissé des pistes : la régulation médicale, la création des services d’accès aux soins (SAS), le renforcement des assistants de régulation, la télémédecine, ou encore une meilleure rémunération des gardes pour les médecins libéraux. Force est de constater que ces solutions ne suffisent pas : elles sont des pansements sur une plaie béante.

t elle eues sur la nature des contrats signés par les hôpitaux pour assurer des gardes complètes ? Alors que le déficit des hôpitaux publics pourrait atteindre 2 milliards d’euros en 2024, quelles mesures comptez vous prendre pour freiner cette spirale onéreuse qui ne permet pas l’accès aux soins pour tous, partout ? En janvier dernier, le Président de la République a exprimé sa volonté de « régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent à bout de bras nos services de soins ». exercent sous un statut d’interne très peu rémunéré. Sans eux, de nombreux services d’urgence ne pourraient plus fonctionner. Ces médecins, essentiels au fonctionnement de nos hôpitaux, vivent dans une précarité tant financière qu’administrative. Ils doivent renouveler chaque année, voire tous les six mois, leur autorisation de séjour, et bénéficient

étudiants français ayant fait leurs études à l’étranger. Il est indispensable de faciliter leurs démarches, afin qu’ils puissent revenir en France faire leurs stages et leur internat, puis exercer. Nous ne pouvons nous permettre de nous priver de leurs compétences. Trop de jeunes choisissent d’étudier la médecine à l’étranger ; cette réalité est alarmante. Madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement envisage t il pour rapatrier les étudiants français formés à l’étranger et même éviter qu’ils ne partent ? Cet été a également révélé l’existence d’un système d’urgences à deux vitesses dans notre pays. Alors que des moyens exceptionnels ont été déployés pour répondre aux besoins sanitaires lors des jeux Olympiques de Paris 2024, les fermetures de services d’urgence se sont multipliées ailleurs en France. Malgré l’afflux massif de touristes en région parisienne pour ce formidable événement, l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP HP) s’est félicitée de la robustesse du dispositif de prise en charge des athlètes et du public. Avec 370 lits supplémentaires ouverts pour la période des Jeux, elle a réussi à fluidifier les passages dans les services d’urgence. réjouissons de ce succès. Il démontre manifestement que lorsqu’une organisation et des moyens adéquats sont déployés, le système fonctionne, et même très bien ! Il est temps de poser un diagnostic clair : notre système de santé est en sursis. Nous devons cesser de le rafistoler avec des solutions à court terme. Il faut une réforme systémique, qui prenne en compte l’ensemble de la chaîne de soins, depuis la prévention et la médecine de ville jusqu’à l’hôpital. Nous devons recréer un maillage territorial cohérent, réhabiliter les services de proximité, redonner aux soignants les moyens de travailler dignement et efficacement. Cette réforme doit se faire en lien avec chaque bassin de vie, en concertation avec les professionnels de santé, les associations de patients et les collectivités locales, qui sont en première ligne pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Pour beaucoup, les urgences sont la porte d’entrée de l’hôpital. Quand elles s’effondrent, c’est tout notre système qui vacille.

régulé au service des urgences dans le département oblige les pompiers et les ambulanciers privés à réaliser des trajets beaucoup trop importants, dans de mauvaises conditions. La prise en charge des patients est indigne. Les médecins intérimaires doivent être réaffectés sur des postes vacants. Les praticiens à diplôme hors Union européenne doivent être régularisés. Nous devons accueillir des brigades cubaines comme pendant la covid 19 dans nos territoires ultramarins, en attendant qu’un nombre suffisant de médecins soit

L’argent doit être au service du bon sens ! » Tout est dit ! Madame la ministre, que répondez vous à Virginie ? Le Gouvernement a t il l’intention de répondre à l’urgence actuelle que connaît l’hôpital public ?

de me donner l’occasion de débattre ce soir de la situation des urgences durant l’été dernier et des perspectives que nous devons emprunter. Vous le savez, j’ai pris mes fonctions il y a quelques semaines, le 21 septembre 2024, c’est à dire le dernier jour de l’été. Je tâcherai néanmoins de répondre à vos questions le plus précisément possible, dans un dialogue que j’espère fructueux. Et je suis bien sûr à votre écoute. Permettez moi dans un premier temps de revenir sur la réalité des tensions qui ont existé cet été au sein des services d’urgence. Quelques chiffres, tout d’abord. La fréquentation des urgences a été relativement stable entre l’été 2024 et le précédent,

Ces chiffres masquent évidemment la grande diversité des situations dans les territoires. Il reste encore des services pour lesquels la période estivale a été source de tensions. Les représentants des urgentistes nous l’ont dit, et vous serez certainement plusieurs ce soir à en faire également

ouverts par la récente réforme des autorisations, ont permis au cas par cas de stabiliser des organisations en s’appuyant sur tous les acteurs du système de santé – je tiens d’ailleurs à souligner ce soir leur grand professionnalisme. Permettez moi également de saluer l’engagement de l’ensemble de la communauté hospitalière, qui s’est organisée pour faire face aux tensions. Je pense évidemment à la mobilisation des médecins des urgences, mais aussi à celle des personnels d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à celle de l’ensemble des soignants et personnels administratifs qui se sont engagés, quitte parfois à reporter,

En 2025 encore, l’Ondam augmentera de 2,8 %, soit 9 milliards d’euros de plus qu’en 2024. y a ensuite une politique d’attractivité des métiers sans précédent. Le Ségur de la santé a marqué une première étape historique pour rémunérer les personnels hospitaliers à la hauteur de leur engagement et susciter des vocations. Nous avons depuis lors engagé la pérennisation des mesures de revalorisation du travail de nuit et du week end, particulièrement importantes quand on exerce aux urgences. En ce qui concerne plus spécifiquement les urgences,

à l’entrée des urgences ou à la réorientation vers la ville des patients ne relevant pas de la médecine d’urgence. Toutes ces mesures, très attendues des acteurs de terrain, sont accompagnées de guides et d’appuis à leur déploiement.

nous organisons le système de santé pour que, à toute heure de la journée, les citoyens puissent accéder à des soins non programmés, après un simple appel téléphonique. Une meilleure organisation de l’accès aux soins permet au bout de la chaîne de soulager les urgences.

pour améliorer l’accès aux soins, qui témoigne des nouvelles relations de confiance et de soutien qui se nouent entre la ville et l’hôpital, ce qui était absolument indispensable.

Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de deux minutes maximum, y compris l’éventuelle réplique. Le Gouvernement dispose pour répondre d’une durée équivalente.

Les services d’urgence, véritables vitrines des établissements hospitaliers, avaient alors décidé de baisser le rideau en nuit profonde à Perpignan. Quel symbole de leur dégradation ! L’été dernier, des personnes ont attendu vingt

n’est pas alarmiste : il s’agit malheureusement d’un cri d’alarme. La réalité des urgences, c’est cet usager qui souhaite passer devant un enfant en situation d’urgence vitale. Ce sont ces familles qui attendent sans information pendant des heures et des heures. Ce sont, encore, ces personnes âgées

que pensez vous faire pour améliorer la régulation des passages aux urgences ? La parole

entre les secteurs public et privé. L’objectif de ce travail sera notamment de redéfinir la répartition des filières de prise en charge de l’aide médicale urgente entre les acteurs.

de ce débat. L’été 2024 a révélé une nouvelle fois la crise des urgences médicales en France, avec non seulement des fermetures perlées, le soir, la nuit et le week end, mais aussi les terribles

En Nouvelle Calédonie, par exemple, nombre d’hôpitaux ont fermé cet été leur service d’urgences la nuit et le week end. Dans plusieurs territoires ultramarins, les problèmes de continuité territoriale affectent l’accès aux soins.

Sous l’impulsion du dernier comité interministériel des outre mer (Ciom), mes prédécesseurs ont lancé des chantiers spécifiques pour retravailler le parcours de santé dans ces territoires. La mesure 23 dudit Ciom vise notamment à fluidifier les prises en charge, particulièrement pour les pathologies lourdes, comme les cancers.

patients. Si la Lozère est relativement épargnée par ce problème, tel n’est pas le cas de certains départements voisins, comme l’Aveyron. Par exemple, à Saint Affrique, l’accès aux urgences de l’hôpital est régulé depuis juin dernier en raison d’un manque de médecins. Dans cet établissement, un seul médecin est en poste pendant vingt pour assurer l’accueil, la gestion des lits de courte durée ainsi que les sorties du service mobile d’urgence et de réanimation (Smur).

Dans les déserts médicaux, bon nombre de professionnels constatent un report de la patientèle dépourvue de médecin traitant vers les services d’urgences pour des soucis de santé qui relèvent plutôt de la « bobologie ». Enfin, les Padhue sont toujours confrontés sont toujours confrontés à des procédures administratives qui compliquent leur intégration dans nos hôpitaux. Madame la ministre, pouvez vous nous indiquer s’il existe une évaluation régulière et qualitative

Les financements de l’assurance maladie pour les activités de psychiatrie ont augmenté de près de 32 % entre 2020 et 2023. Ils atteignent désormais 12 milliards d’euros

proposer trois formes de prise en charge : des séjours à temps complet, des séjours à temps partiel et des soins ambulatoires. Cette réforme prévoit également un fonctionnement en réseau,

les gouvernements se déclarent satisfaits quand « seulement » 46 % des établissements ferment leurs services durant la période estivale. Pour les élus locaux, les mois de juillet et d’août sont au contraire source de tensions et d’angoisses.

Allez vous déployer les moyens nécessaires le prochain projet est à Mme la ministre. Madame la sénatrice, le centre hospitalier de Briey rencontre des difficultés de recrutement depuis plusieurs années,

pu résoudre les problèmes posés à sa ligne de garde, il a fait le choix de maintenir l’organisation validée et communiquée aux parturientes, afin d’éviter toute confusion. Cet établissement bénéficie d’un suivi resserré des équipes de l’ARS.

sociales (Igas), la permanence des soins en établissement était assumée à 82 % par les hôpitaux publics, quand le secteur privé n’en assurait que 13 %. De plus, seuls 39,34 % des médecins libéraux participaient à la permanence des soins ambulatoires.

La dernière étude annuelle de l’ordre des médecins sur la permanence des soins ambulatoires indique que 39 % des médecins généralistes ont participé à la permanence des soins en 2023 – vous l’avez rappelé vous même. un total de 66 257 médecins susceptibles de prendre une garde. Un médecin réalise en moyenne vingt huit gardes chaque année et l’âge moyen des effecteurs de gardes est de 45 ans.

Madame la ministre, la population et les élus des territoires vous demandent d’agir efficacement. Nous n’attendons pas de miracle : nous exigeons simplement ce qui est dû. Comment comprendre que les cliniques privées refusent de prendre en charge certains actes jugés non lucratifs, les renvoyant aux urgences de l’hôpital public ? Comment comprendre que les groupements hospitaliers de territoires (GHT) en soient réduits à gérer des pénuries par un système de reconcentration des moyens autour des métropoles, alors qu’ils devaient servir de leviers de bonne répartition des moyens sur l’ensemble du territoire

M. Daniel Chasseing. Madame la ministre, pendant l’été 2024, la situation des urgences a été difficile dans de nombreux territoires, notamment

qui ont été très solidaires et très professionnels. Ces fermetures et difficultés sont dues à un manque de médecins urgentistes, à des tensions sur le personnel et à une hausse de

généraliser le triage à l’entrée, afin que les urgences mineures soient prises en charge dans une salle différente par un médecin généraliste ; deuxièmement, disposer

aussi, madame la ministre,

demeurent insuffisants pour répondre à la demande croissante des patients. Cette pénurie se traduit par un engorgement des services d’urgences, par des conditions de travail de plus en plus difficiles et par une fatigue accrue des équipes. En somme, nous sommes toujours face à une situation critique. En 2020, par exemple, 77 % des structures d’urgences étaient publiques. Elles ont pris en charge 18 millions de passages, même si l’on a observé une baisse de 17 % par rapport à l’année précédente, en raison notamment de la pandémie. Au fil des années, les problèmes persistent. Le manque de ressources, tant humaines que matérielles, maintient les services d’urgences dans une crise permanente. Pour tenter de limiter l’afflux, des mesures de régulation ont été instaurées. Celles ci, bien que nécessaires, sont souvent mal perçues par les patients et engendrent de l’incompréhension.

d’accueillir, d’évaluer rapidement le degré d’urgence et d’organiser le début du parcours dans une structure adaptée aux besoins du patient.

Cet été, le service d’urgences de cet établissement clé pour notre territoire a dû régulièrement fonctionner de nuit avec quatre urgentistes, alors que six sont nécessaires. Par ailleurs, la fermeture régulière des services d’urgences d’autres hôpitaux situés à proximité, comme ceux de Digne les Bains et de Manosque, a provoqué des reports vers l’hôpital d’Aix,

dont le dévouement a pour limite leur capacité physique à supporter une charge de travail toujours plus lourde. Il devient d’ailleurs de plus en plus difficile de recruter dans certaines

la crise politique a de graves conséquences sanitaires. Il a été difficile, voire impossible, d’accéder au centre hospitalier territorial, en raison des barrages. Depuis le 2 septembre dernier, les lits d’hospitalisation sont fermés à Poindimié et à Koumac, faute d’infirmiers et de médecins. Il n’y a plus eu de services d’urgences de nuit durant de nombreuses semaines, et peut être est ce encore le cas aujourd’hui. Le nombre de décès a presque doublé. Permettez moi d’évoquer les problèmes que nous avons connus à La Réunion, non pas cet été, mais durant notre hiver austral.

Il s’agit, mes chers collègues, vous qui représentez les collectivités territoriales, de l’ancien maire de Salazie, Jean Claude Welmant. Vous en conviendrez, une si longue attente est inacceptable pour tout citoyen, ancien maire ou non. Cette grave défaillance reflète la situation fragile de notre CHU, et ce malgré l’engagement remarquable des équipes. Au delà des spécificités liées à l’insularité, le service des urgences du CHU de La Réunion,

C’est l’honneur de notre CHU, c’est l’honneur de La Réunion, mais il y va aussi de l’image de la France dans son bassin régional. Cela suppose toutefois un soutien de l’État. Le précédent gouvernement avait annoncé une revalorisation de trois points du coefficient géographique, ce que l’ensemble des acteurs avaient accueilli avec satisfaction.

avoir une pensée pour tous ceux qui œuvrent en faveur de l’apaisement, notamment nos forces de l’ordre, les fonctionnaires de l’État, mais aussi les responsables politiques et syndicaux ainsi que les acteurs de la société civile, qu’ils soient issus du monde économique, religieux ou coutumier.

Je suis consciente des contraintes spécifiques, que vous avez décrites, auxquelles cet établissement est confronté, sans oublier l’éloignement géographique, les surcoûts logistiques et la forte demande de soins, dans un contexte sanitaire plus complexe que celui de l’Hexagone.

Ce soutien financier important va de pair avec un travail mené par la gouvernance du CHU sur le fonctionnement de l’établissement et la fluidité des parcours. Vous évoquez le coefficient géographique, rehaussé de 31 % à 34 %. Cette réévaluation s’applique sur les tarifs et

Mes prédécesseurs s’y sont engagés et je m’inscris dans cette approche : nous devons aider le territoire mahorais à se doter de leviers d’attractivité et de fidélisation de ses professionnels de santé.

Le dimanche, un proche atteste que la personne était totalement incapable de se déplacer, de s’alimenter et de satisfaire à ses besoins naturels – deuxième manquement grave au service public de la santé. Le lundi, nouvelle hospitalisation en urgence, cette fois à Auch, où est diagnostiquée une grave infection, avec insuffisance pulmonaire et prescription de dialyse tous les deux jours.

du sud de l’Alsace, région où trois frontières s’entremêlent, ce qui complique encore la situation dans laquelle se trouve notre système de soins. Dans ce territoire, comme partout ailleurs, une frange importante de la population est vieillissante et les maladies chroniques sont en constante augmentation. Comme ailleurs encore, la médecine de ville est carencée. Les listes d’attente chez les rares spécialistes s’allongent, décourageant bon nombre d’habitants qui finissent par renoncer à se faire soigner. Dans les hôpitaux du sud de l’Alsace, les urgences peinent à accueillir des patients qui se présentent régulièrement, faute de trouver à se soigner ailleurs dans la durée. Je pense tout particulièrement aux personnes âgées, notamment aux plus isolées Dans le secteur des trois frontières, le phénomène d’aspiration des personnels de santé vers les pays voisins aggrave encore les choses : chaque jour, 250 soignants traversent le Rhin pour travailler en Allemagne

francs suisses bruts par mois, mais aussi qualitatives, en raison de meilleures conditions de travail et de formation. L’hôpital de Saint Louis, à quelques mètres de la frontière, est à cet égard particulièrement affecté. La Collectivité européenne d’Alsace a mis en place une politique spécifique pour valoriser ce secteur géographique, le rendre plus attractif et favoriser l’installation des personnels de santé. Toutefois, dans un contexte de forte concurrence entre les territoires, les capacités de cette collectivité atteignent leurs limites. Alors que des leviers ont été identifiés pour limiter les conséquences de ce phénomène de fuite, comment le Gouvernement compte t il rendre effectives les conventions de coopération sanitaire, notamment celles de 2016, pour répondre aux besoins particuliers de ce territoire ? La parole est à Mme

mais il y va de l’intérêt des Suisses et des Français habitant de part et d’autre de cette frontière. Les données de l’Observatoire statistique transfrontalier (OST) mettent en évidence un important déséquilibre entre le lieu de résidence et le lieu de travail des soignants exerçant en Suisse.

De crise en crise et de plan blanc en dispositif provisoire, la vision court termiste des services hospitaliers nous conduit à un échec certain et mortifère.

Ces mots sont ceux d’un soignant cité dans l’enquête de Samu Urgences de France, publiée le 17 septembre dernier : ils doivent nous alerter. La situation des urgences dans notre pays est préoccupante. Ce débat, proposé par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, a été l’occasion pour nous tous d’exprimer notre inquiétude, notre colère aussi, face à une situation qui se répète chaque année au grand dam de nos concitoyens. concitoyens. L’hôpital brûle et, malgré les promesses, rien ne change. Les chiffres évoqués ce soir sont éloquents deux services d’urgences sur trois ont fermé au moins une fois cet été ; un tiers ont dû mettre en place une régulation médicale d’accès par le 15 ; quatre vingt six départements ont été touchés par la fermeture d’au moins une ligne médicale. Si le bilan est meilleur qu’en 2023, il convient de l’analyser au regard du nombre anormalement élevé d’heures supplémentaires. Le personnel tient au prix d’un sacrifice trop peu reconnu. Malgré la crise, 1 500 lits ont été fermés et près de 1 000 postes d’internes ont été supprimés en 2024 – une aberration En métropole comme dans les territoires d’outre mer, les urgences ne sont plus en mesure de mener à bien leurs missions. Dans le département dont je suis élu, la Dordogne, les urgences de l’hôpital de Sarlat ont dû fermer plusieurs jours consécutifs cet été

départementaux d’incendie et de secours qui assurent les transports, notamment des sapeurs pompiers volontaires, pourtant libérés par leurs employeurs pour participer aux opérations de secours et non pour pallier les carences de notre système de santé.

Les mesures passées sont insuffisantes, les quelques effets positifs de la mission flash de 2022 ne sont pas à la hauteur, la désorganisation et les dysfonctionnements de notre système de santé sont beaucoup trop profonds. Face à cet effondrement, des structures privées émergent et permettent de compléter l’offre de soins. Centres médicaux privés ou cabinets à horaires élargis proposent une prise en charge des petites urgences. Ils se veulent l’échelon manquant entre urgences et généralistes. Cependant, ils ne peuvent se substituer à l’hôpital public. Mes chers collègues, l’égalité d’accès aux soins est l’une des bases de notre système de santé. Nous ne pouvons laisser s’imposer une médecine à deux vitesses. Des lits et des bras ! », voilà ce que réclament les soignants pour sauver les services d’urgences. Leur mission première est de soigner, de sauver des vies, et ils doivent pouvoir le faire dans de meilleures conditions. Nous nous faisons le relais des propositions formulées par Samu Urgences de France.

Les services d’urgences ne peuvent plus répondre aux besoins croissants de la population. Revoir le maillage territorial des services d’accueil est donc une nécessité. Il nous faut plus de centres de soins primaires ; nous devons également généraliser progressivement la régulation médicale d’accès aux urgences

de psychiatres et de psychologues. En ce domaine, nous ne sommes pas à la hauteur des besoins : il est urgent d’agir vite et bien pour répondre présent face à la demande croissante.

Les élus sont en première ligne : certains, en Bretagne et dans le Sud Est, ont même pris des arrêtés appelant à un plan d’urgence d’accès à la santé.